et favorise les importations, ce qui dégrade notre empreinte environnementale et réduit notre capacité à atteindre les objectifs de la stratégie bas-carbone. C'est bien par la souveraineté alimentaire que nous maîtriserons mieux le bilan carbone de notre alimentation

l'étude, nous amène à nous pencher sur notre alimentation, en engageant une transformation de nos habitudes vers un modèle plus responsable. Notre façon de nous alimenter constitue en effet un levier non négligeable de lutte contre le réchauffement climatique. Au sein de ce volet, l'article 59, relatif au menu végétarien dans la restauration collective, revêt une importance particulière. En effet, on estime à 30 % la réduction des émissions de gaz à effet de serre susceptible de résulter du remplacement d'un menu non végétarien par un menu Aussi, je regrette que la commission soit revenue en partie sur cet article et qu'elle ait privilégié une prolongation de deux ans de l'expérimentation introduite par la loi Égalim, au détriment de sa généralisation. Il s'agit, selon moi, d'une régression par rapport à la proposition initiale, qui était pourtant équilibrée. L'objectif est avant tout de garantir aux élèves un accès à une liberté de choix et à une alimentation saine, plus locale

dans les cantines démontre que ces menus sont plutôt bien entrés dans les habitudes et que la plupart des réserves à ce sujet ont été surmontées. L'expérimentation a démontré qu'il est possible de permettre à chacun de quand il le souhaite, de la viande, et de la viande de qualité, mais également qu'il est possible de diversifier ses apports de protéines, sans pour autant stigmatiser la consommation de viande. Il faut conclure,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 59 de ce projet de loi prévoit l'instauration, à titre expérimental, d'un repas végétarien au moins une fois par semaine dans les services de restauration collective scolaire. Avant même que nous ne débattions plus concrètement de cet article, je souhaite souligner deux points forts, qui font écho aux nombreux débats et aux fausses polémiques relatifs aux menus végétariens. Les opposants à cette expérimentation mettent souvent en avant l'impossibilité de mettre en place ces repas dans les services de restauration collective ou encore la ferme opposition des éleveurs. premier lieu- je pense que nous pouvons tous en faire l'expérience, chacun dans notre territoire -, de nombreuses collectivités ont déjà instauré des menus végétariens, selon des rythmes qui varient, au sein de leurs structures de restauration collective. Simplement- c'est du bon sens et non du dogmatisme, comme on peut parfois l'entendre il a bien entendu fallu un temps d'adaptation ; mais rien n'est insurmontable. En deuxième lieu, cessons d'entretenir cette opposition stérile entre les éleveurs et l'instauration d'un seul repas végétarien hebdomadaire. Les éleveurs et les producteurs de viande, dont je fais partie, ont bien conscience de la nécessité de changer, au moins modestement, notre production et notre consommation.

faire le choix de la qualité de notre viande, c'est évidemment favoriser la production locale, dans nos territoires et, ainsi, avoir un meilleur bilan environnemental par rapport à de la viande importée, à tous points

également l'Europe -dépendons des protéines végétales sud-américaines ; nous importons du soja brésilien pour la consommation de notre bétail ou pour la consommation humaine. Il nous faut absolument sortir de cette dépendance, parce qu'importer des protéines végétales

l'équipe pédagogique et administrative des collèges et des lycées continue de dépendre du ministère de l'éducation nationale ; il y a donc une bigouvernance, puisque certains agents relèvent des collectivités et d'autres du ministère de l'éducation Le fonctionnement du service de restauration dépend de la bonne collaboration entre l'équipe de cuisine, dont le chef de cuisine, qui dépend du département ou de la région, et le gestionnaire de l'établissement lui-même, qui se trouve sous l'autorité du proviseur, lequel dépend du ministère de l'éducation si les collectivités attribuent bien le budget de restauration collective aux gestionnaires, ce sont ces derniers qui sont ensuite chargés des dépenses et de la facturation des achats de biens et de services de tout l'établissement, avec une autonomie dans les choix budgétaires, dans le cadre de cette enveloppe. C'est pourquoi la composition et la qualité des menus peuvent différer, sur le terrain, entre deux établissements scolaires pourtant voisins. Cela signifie que les départements et les régions qui seraient volontaires pour participer à cette expérimentation

celle des collectivités. Ainsi, au nom de l'exemplarité de l'État dans la transition écologique, il faut permettre aux collégiens et aux lycéens d'avoir le choix, dès lors que plusieurs plats sont proposés.

expérimentation sera proposée dans un autre article du projet de loi, qui permet de disposer des données évaluatives sur le sujet. Enfin, pour éclairer les débats, je signale que l'amendement que nous examinons supprime la possibilité d'un choix de menus végétariens quotidiens dans les restaurants collectifs du personnel des collectivités territoriales volontaires

succès, malgré une faible anticipation de la part de certaines collectivités et en dépit d'un contexte sanitaire complexe. C'est le succès démontré par cette étude qui a conduit les députés à adopter cette mesure.

peut permettre à ces collectivités d'avancer sur le sujet. Or cet accompagnement a précisément été inscrit dans le présent projet de loi, qui prévoit la définition, par l'État, d'outils d'aide à la décision, à la structuration des filières, à la formulation des marchés publics

Si la mise en place de cette mesure nécessite une phase de transition déjà amorcée, elle est bénéfique pour les collectivités, les usagers et les territoires ; le repas végétarien hebdomadaire permet de s'appuyer sur des menus à base de protéines végétales moins coûteuses

Cet amendement de repli vise à généraliser l'expérimentation d'un menu végétarien hebdomadaire tout en excluant, jusqu'en 2025, les restaurants servant moins de 200 couverts par jour. En effet, les données et les retours des acteurs de terrain montrent que ce sont principalement les collectivités concernées par de petits services de restauration collective qui ont eu des difficultés à mettre en oeuvre cette mesure. Ainsi le sondage de l'AMF, sur lequel s'est fondée la commission des affaires économiques pour revenir sur la généralisation de l'expérimentation,

puissent s'approprier ces questions. Les textes budgétaires ont amorcé un soutien à la transition- nous l'avions sollicité depuis des années -qu'il est important de renforcer. Il s'agit également de prendre en compte les réalités différenciées des collectivités, tout en maintenant le cap clair le cap clair de la transition vers une diversification des sources de protéines. Cet amendement vise donc, afin de trouver un compromis, à accorder un délai supplémentaire de deux ans aux petites villes en généralisant l'expérimentation pour les restaurants collectifs de plus de 200 couverts, et en reportant l'entrée en vigueur de cette mesure à 2025 pour les petits restaurants. Je le répète, le repas végétarien hebdomadaire, après une période de transition qui peut induire temporairement de la complexité est,, bénéfique bénéfique sur tous les plans. Il permet de répondre à la demande. Cela ne signifie pas se détourner de la viande, mais en manger moins pour se tourner vers de la viande de qualité et locale. Moins

On le sait, pour réussir la transition agroécologique, il faut allonger et diversifier les rotations et cultiver des légumineuses qui fixent l'azote dans le sol.

Face à une montée en puissance des modes de vie végane, végétarien et végétalien, il est impératif que les établissements scolaires continuent de proposer des plats à base de protéine animale aux nombreux écoliers, collégiens et lycéens que compte notre pays.

Cette évaluation doit tenir compte de l'impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas. Toutefois, nous estimons qu'un aspect très important est actuellement occulté, celui de la capacité des gestionnaires de s'approvisionner localement. La demande sociétale en matière de circuits courts est de plus en plus forte, nous pouvons nous en féliciter. Nous appelons de nos voeux une relocalisation de nos productions agricoles et estimons que la restauration collective peut constituer, à cet égard, un levier essentiel.

L'objet de cet amendement est donc de prévoir que l'expérimentation de l'évaluation visée à l'article 59 se penche spécifiquement sur la proportion ou le taux d'approvisionnement en produits locaux ou français. L'amendement n° 1106, présenté

L'accès à l'alimentation végétarienne pour nos enfants, synonyme d'une diversification des repas et d'une réduction de l'impact environnemental de l'alimentation collective scolaire, doit être mis en place avec une haute exigence de qualité globale. qualité globale. Cet amendement vise à la fois à offrir un choix et à garantir une qualité. C'est pourquoi nous proposons que l'évaluation de l'expérimentation sur les menus végétariens, prévue à l'article 59, outre le outre le gaspillage alimentaire, la fréquentation et le coût des repas, aborde également la qualité globale des menus, en incluant leur origine, le caractère transformé des produits servis et la consommation d'additifs, colorants ou stabilisants alimentaires. Encore une fois, cet amendement concerne en premier lieu l'expérimentation du menu végétarien, mais vise l'objectif d'étendre, au fond, le principe à une qualité d'ensemble pour la totalité des repas servis. L'amendement

et privée en 2024. Il convient, dès maintenant, d'acter le principe de sa généralisation au-delà de la seule restauration scolaire, afin de créer durablement des débouchés locaux pour une viande de qualité et pour la structuration des filières de protéines végétales à destination de l'alimentation humaine. On ne le répétera jamais assez, aujourd'hui, la majeure partie de la viande en restauration collective est encore issue d'importations. Il est donc nécessaire de développer la demande pour une viande locale de qualité et produite dans le respect de l'environnement. L'introduction de protéines végétales en restauration collective est un levier pour atteindre cet objectif d'approvisionnement en viande locale et de qualité. Les faits démontrent les restaurants collectifs qui pratiquent le plus les repas végétariens sont ceux qui servent de la viande issue de circuits de proximité et de pratiques de production durables. Il s'agit également de rendre cette viande de qualité accessible au plus grand nombre, ces restaurants collectifs. De même, afin de réduire la fertilisation azotée et de développer une alimentation moins émettrice en gaz à effet de serre, il est nécessaire de développer les cultures de légumineuses, y compris pour l'alimentation humaine. Le Gouvernement, la stratégie nationale sur les protéines végétales, cherche à engager la France dans le développement de productions légumineuses- c'est extrêmement louable -, notamment en légumes secs. Pour ce faire, des filières sont encore à structurer et des débouchés à construire. La restauration collective peut jouer un rôle

proposent quotidiennement le choix d'un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. » Je ne saisis pas l'utilité de cet ajout, si ce n'est d'établir et de voter des lois totalement bavardes et inutiles, dont les collectivités ne sauront que faire.

nous proposons que la mise en place d'une option végétarienne, prévue par le présent projet de loi pour les restaurants collectifs gérés par l'État, soit étendue à toute la restauration collective en 2025.

issue de nos systèmes d'élevage durables et familiaux, caractérisés notamment par une alimentation à l'herbe des animaux- 80 % en ce qui concerne le cheptel allaitant -et une autonomie alimentaire du troupeau ». La relocalisation de la qualité de l'offre de viande proposée en restauration collective est essentielle pour l'environnement et le revenu des éleveurs. Les pratiques de terrain confirment cette analyse : les restaurants qui proposent des menus végétariens sont aussi ceux qui travaillent à un approvisionnement en viande locale et de qualité. Alors que, aujourd'hui, 38 % des Français se disent flexitariens, la grande majorité d'entre eux, soit 96 %, achète toujours de la viande, mais de meilleure qualité. N'opposons surtout pas protéines végétales et viande, bien au contraire ! Une option végétarienne quotidienne s'inscrit donc dans cette évolution de la demande sociétale du « manger moins et mieux » de viande, pour ceux qui mangent de la viande, afin de préserver l'environnement et de privilégier l'économie locale et de qualité. La mesure

qui n'ont pas les moyens de proposer deux menus. De plus, elle entrerait en vigueur en 2025, pour laisser le temps de la transition aux acteurs. L'amendement n° 2055, présenté

L'article 59 vise à prévoir la création d'une expérimentation pour les collectivités volontaires leur ouvrant la possibilité de proposer, dans les services de restauration collective dont elles ont la charge, le choix d'un menu végétarien quotidien. Il indique également, dans son alinéa 5, que les collectivités volontaires font connaître au représentant de l'État dans le département leur engagement dans l'expérimentation, afin d'en faciliter l'évaluation. Toutefois, il apparaît que l'échelon régional est le plus pertinent pour assurer ce rôle de recensement. En effet, ce sont les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (Draaf) et les directions de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts (Daaf) qui examinent la déclinaison territoriale de la politique d'alimentation. À ce titre, pour des raisons de coordination territoriale, cet amendement vise à confier ce recensement à l'échelon régional et non départemental. n° 279 rectifié. La formulation actuelle de l'article 59 peut semer le doute chez les acteurs de terrain de la restauration collective. En effet, il n'est pas expressément dit que les structures relevant de la responsabilité de l'État, mais faisant appel à un prestataire de services pour préparer tout ou partie des repas, sont concernées par l'article. Pourtant, c'est le cas d'une grande partie de ces structures. Il est donc important d'être plus explicite dans la rédaction de cet alinéa afin d'en améliorer, ensuite, son appropriation.

l'organisation d'une concertation tout au long de l'expérimentation afin de veiller au bon déploiement de celle-ci. Elle associera les collectivités territoriales ainsi que leurs regroupements et le représentant de l'État dans la région. Or la loi Égalim a créé des comités régionaux pour l'alimentation (Cralim), dont le rôle est la mise en oeuvre, au niveau régional, du Programme national pour l'alimentation et notamment la déclinaison des politiques publiques en restauration en restauration collective. À ce titre, nous proposons que la concertation prévue par cet article soit réalisée au sein de ces mêmes comités régionaux. Cela permettrait d'éviter la création d'une nouvelle instance de concertation uniquement consacrée au suivi de l'expérimentation et de s'inscrire en pleine cohérence avec les dispositions de la loi Égalim.

de prévoir, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson et composé de protéines animales ou végétales. Si nous voulons être efficaces, il faut cibler l'ensemble de la restauration collective. Pourquoi exonérer de ces objectifs les restaurants collectifs et cantines des personnes morales de droit privé ? Les deux amendements

des apports en protéines dans notre alimentation. Il semble en effet normal que la restauration collective privée, au même titre que les collectivités, permette à chacun de choisir son alimentation. Encore une fois, il ne s'agit pas de stigmatiser la consommation de viande ou, encore moins, nos éleveurs, mais plutôt de privilégier une alimentation de qualité. Une augmentation de la part de protéines végétales dans notre alimentation contribuerait, on le sait, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'au renforcement de notre souveraineté alimentaire. Cet amendement vise

donc que les crèches soient concernées de la même façon que les cantines scolaires. besoins des usagers, les crèches gérées par des personnes morales de droit public ou privé sont tenues de permettre, y compris sur inscription, une option sans viande ni poisson à chaque repas, composée en majorité de protéines végétales.

1900 et 2058.

soit en voulant aller plus loin, soit en voulant revenir en arrière. Il s'agit des amendements n 275 2175, 1896, 1897, 1370

La commission ne souhaite pas revenir sur les engagements pris dans la loi Égalim auprès des acteurs concernés et tient à respecter le calendrier issu du travail parlementaire. Comment peut-on demander à des parlementaires de généraliser une expérimentation, sans s'appuyer sur une évaluation fiable de la mesure ? Certes, un rapport a été remis, monsieur le ministre, mais il est partiel et, finalement, admet clairement qu'il est impossible de conclure. Je vous en citerai un certain nombre de passages. Au départ, le dispositif s'est heurté à des réticences et a confronté les opérateurs à de grandes difficultés pratiques. Ensuite,

La notion même d'expérimentation suppose de partir d'un point 0 clairement identifié et de se fixer des indicateurs. Le calendrier de mise en oeuvre de la mesure ne l'a pas vraiment permis. Les inspecteurs ajoutent « regretter de ne pas disposer encore de chiffres exhaustifs et fiables rendant compte avec précision de la réalisation de l'expérience ». Le rapport devait mesurer l'impact de l'expérimentation sur le coût du repas, la fréquentation et le gaspillage alimentaire. Sur ces thématiques, « l'impact de la mesure sur la fréquentation la date de production du rapport par manque de données chiffrées ». « L'impact de la mesure sur le prix de revient des repas n'a pas non plus pu être établi de façon précise [ ...] par manque de données chiffrées. » « L'impact de la mesure sur le gaspillage alimentaire n'a pas non plus pu être établi de façon précise.

savoureux ». Tout cela les amène à conclure qu'il est utile non pas de pérenniser, mais bien de mener l'expérimentation à son terme et de stabiliser la situation sans s'interdire de la faire évoluer. dès lors incontestable qu'il n'est, aujourd'hui, pas possible de tirer un quelconque enseignement des deux années passées d'expérimentation d'un menu végétarien hebdomadaire en restauration scolaire, globalement en raison de la crise du C'est sans doute pourquoi 75 % des maires interrogés s'opposent à cette pérennisation et pourquoi, monsieur le ministre, votre majorité demande, à l'amendement n° 2064, le report

La commission déplore cette pratique qui consiste à proposer des expérimentations d'une durée courte puis, sans évaluation, à les généraliser après à peine un an.

La commission des affaires économiques propose donc une solution de sagesse sur ces menus végétariens : non pas une pérennisation d'une expérimentation sans évaluation, mais une prolongation prolongation de deux années supplémentaires, qui compenseront les dix-huit mois de période covid-19 et permettront de disposer du recul nécessaire pour une véritable évaluation. Il y va, monsieur le ministre, mes chers collègues, de l'objectivité de cette démarche. Cette option permettra aux élus locaux ayant déployé des efforts importants pour mettre en place ces menus de continuer d'en mesurer les effets. Pour d'autres, elle permettra de poursuivre, voire, pour les plus volontaires, de coup d'arrêt dans le déploiement des repas végétariens pour les volontaires. Pendant ce temps, chose importante, nous pourrons consolider nos capacités d'approvisionnement en produits locaux et français.

La seconde question est celle de savoir s'il faut aller plus loin, avec plus d'un menu végétarien par semaine en restauration scolaire ou un menu par semaine dans les crèches. À ce également, il me semble essentiel de soutenir la position d'équilibre de la commission. Je le rappelle, d'un point de vue nutritionnel, l'Anses s'estime incapable de trancher la question de la qualité nutritionnelle de plus d'un menu végétarien par semaine

À ce stade, il me paraît inutile de préciser dans la loi une obligation pour les self-services des personnels privés, dans la mesure où cette restauration pratique déjà l'offre végétarienne, souvent bien au-delà d'un menu par semaine.

des collèges et des lycées. Voilà ce qu'il faut encourager !

ont adoré et en redemandent ! Cette opération a permis à des enfants qui n'ont pas forcément l'occasion de manger du gibier à la maison de découvrir des produits nouveaux, de manière ludique. C'est un partenariat gagnant-gagnant avec la collectivité, la fédération des chasseurs et la chambre d'agriculture qui permet de développer des filières locales, de proposer de la viande de qualité et de faire face à la surpopulation de gibier, dont on connaît les dégâts pour le monde agricole. La CEA a donc proposé cette viande en circuit court et en proximité dans les collèges et les Ehpad. Ce fut une réussite que je tenais à saluer. Cette initiative départementale montre que, sur le terrain, nous sommes bien loin du dogmatisme qui prévaut chez certains sur ce sujet. Il faut bien évidemment proposer des menus végétariens, mais il convient également d'offrir des repas avec de la viande de qualité issue des filières locales. filières locales. Cela est bénéfique pour tout le monde et fortement apprécié des enfants. Ne légiférons pas sur tout, ni sur le contenu du menu ni sur le diamètre de l'assiette ou la longueur de la fourchette ! Faisons tout simplement confiance aux acteurs locaux de nos territoires.

sénateur varie ... Nous passons notre temps à regretter les obligations que nous imposons aux collectivités et aujourd'hui nous jugerions de la vertu des repas ? Je voudrais saluer la sagesse et la pertinence de la position de la commission des affaires économiques et de sa rapporteure.

relatif aux pratiques dites « de dégagement », qui concernent certains produits alimentaires, notamment le lait, la volaille, le porc ou le boeuf. Plutôt que de stocker ces produits ou de les écouler sur les marchés habituels à des prix très bas, certains opérateurs métropolitains préfèrent les « dégager », c'est-à-dire s'en débarrasser vers les départements d'outre-mer, où ils peuvent notamment servir à fournir les services de restauration collective.

en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. Cet amendement vise donc à en limiter le recours pour les services de restauration collective dans les départements et régions d'outre-mer. Quel est

et, en cas d'échec, de fixer par arrêté l'intensité et la durée des périodes de mise à la distribution des produits de dégagement. Une circulaire de mai 2017 a précisé ces dispositions. Dans son avis de juillet 2019, à la suite d'une saisine du ministre de l'économie, l'Autorité de la concurrence a considéré que, les produits n'étant pas similaires, la situation ne pouvait pas être assimilée à une concurrence déloyale. Elle a formulé à ce titre des recommandations sur le développement des produits sous signes de qualité et sur la structuration des filières. Cette démarche de lutte contre les marchés de dégagement est largement engagée dans certains territoires ultramarins. Je pense

le recours aux produits transformés. Dans un magasin bio, par exemple, un produit sur quatre environ est ultratransformé. Le travail d'élaboration du décret réalisé en bonne intelligence avec les professionnels de terrain permettra d'établir la liste des produits dits « ultratransformés » et facilement identifiables par les gestionnaires des cantines concernées.

des effets préjudiciables sur la santé. Ils sont notamment à l'origine des phénomènes d'obésité, que nous connaissons de plus en plus dans notre pays, et d'allergies, voire plus grave. Je ne considère pas cette mesure comme une punition. Au contraire, c'est plutôt vertueux à tous les niveaux, car nous avons un crucial problème de santé. Pour terminer, je dirai que, dans un pays où le repas gastronomique est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, on se doit d'éduquer au goût et de bannir ce genre de plats.

émis un avis défavorable

Les auteurs de cet amendement pensent qu'il est nécessaire de préciser que l'apprentissage de l'importance des protéines végétales dans l'alimentation humaine au sein des formations initiales et continues relatives à la cuisine doit comporter un aspect pratique et technique de la préparation des légumineuses et autres protéines végétales en plat principal. Vous le savez, monsieur le ministre, l'élevage intensif évoqué par mon collègue Daniel Salmon constitue une part importante des des sources de gaz à effet de serre, notre collègue Ronan Dantec l'a rappelé. Aussi, pour la santé des citoyens et dans le cadre de la lutte contre le dérèglement climatique, qui fait l'objet de cette loi, il nous paraît important de diversifier notre alimentation et, plus précisément, les sources de protéines. Les protéines animales ne sont pas indispensables, nous le savons tous. Pour autant, elles ne doivent pas être supprimées. Toutefois, il convient de tenir compte de leur surconsommation et de ses effets nocifs sur la santé. Le programme Le programme national nutrition santé, le PNNS, établi par le ministère chargé de la santé, recommande le seuil de 500 grammes de viande cuite hors volailles par semaine, alors que, vous le savez parfaitement, notre consommation moyenne en viande est encore nettement au-dessus de ce seuil. Aussi, malgré les polémiques que j'estime injustifiées sur les menus végétariens, l'amendement que nous proposons ici vise à inscrire dans la loi l'obligation, au-delà de ce qui est déjà fait en termes d'apprentissage théorique sur la nécessité de diversifier les sources de protéines, de prévoir l'apprentissage de l'élaboration de plats à base de protéines qui ne sont pas issues d'animaux, de manière pratique et concrète. Le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, que j'ai interrogé sur le sujet des formations de BEP et de CAP, dans le cadre d'une question écrite sur les formations, m'a m'assuré qu'il est « important de noter que les compétences nécessaires à l'élaboration d'une alimentation végétale sont d'ores et déjà intégrées au référentiel définissant les diplômes professionnels de restauration vous pouvez le vérifier sur le site du ministère de l'éducation nationale -, le programme enseigné est encore celui qui est validé par l'arrêté du 17 mars 2016, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte des avancées de la loi Égalim votée en 2018.

Apprendre à cuisiner des protéines végétales en plat principal nécessite d'être mentionné, sans quoi seuls les modules transversaux santé et environnement pourraient intégrer les référentiels. Les cuisiniers pourraient donc être sensibilisés aux avantages théoriques d'une diversification de protéines, mais sans être formés pratiquement et techniquement à la préparation de tels plats. Quel est l'avis de la commission

Il visait ainsi à permettre la modulation de ses tarifs, en fonction d'un barème progressif dont les tranches résultaient de l'application du quotient familial. Il confirmait la possibilité, pour les collectivités ou les établissements gestionnaires, de décider de la gratuité du service de la restauration scolaire pour les plus modestes.

Des différences territoriales fortes demeurent, alors que la précarité est bien présente sur le territoire. Nous sommes nous aussi attachés au principe de libre administration des collectivités

l'amendement n° 1901. L'exigence de qualité nutritionnelle des repas proposés dans le cadre de la restauration scolaire doit bénéficier à tous les enfants, quels que soient leur lieu de résidence et les moyens financiers de leur famille.

L'article prévoyait en outre la possibilité pour les collectivités de déterminer la gratuité de ces repas, selon des modalités de calculs. Nous aurions donc, au lendemain de l'adoption de cette loi, des collectivités qui devraient suivre les modèles déterminés par Paris

méprisent la qualité de l'alimentation. Le quotient familial, c'est la justice ! Les ménages modestes méritent de pouvoir nourrir leur famille correctement. Très souvent, pour les enfants, le repas au restaurant scolaire est leur seul repas équilibré de la journée.

est ainsi libellé : La parole est à M. Henri Cabanel. Introduit par l'Assemblée nationale, l'article 59 du projet de loi propose de lancer une expérimentation visant à mettre en place une solution de réservation de repas dans la restauration collective publique. telle mesure est bienvenue, puisqu'elle permettrait d'adapter l'offre de repas à la demande et de lutter ainsi contre le gaspillage alimentaire. Comme on peut le lire dans le rapport de la commission des affaires économiques, l'expérimentation est ici superfétatoire. Plus nous proposons d'options dans le cadre de la restauration collective, plus le risque est réel pour le gestionnaire de commander des repas qui seront finalement jetés. Dans la perspective de la généralisation à terme des menus végétariens quotidiens, nous considérons que la mesure d'une solution de réservation va de soi. Quel est l'avis de la commission

pour bien évaluer les conséquences d'une telle mesure, les expérimentations trop courtes ne permettant pas de disposer du recul nécessaire. La transformation de l'expérimentation proposée par l'article 59 en obligation me semble donc prématurée à ce stade. Elle constituerait une contrainte,

La première pose comme priorité absolue le fait de tendre vers un maximum de produits sous labels en restauration collective, d'une part, en affichant des objectifs très ambitieux, mais malheureusement peu réalistes au regard des approvisionnements actuels, et, d'autre part, en restreignant la liste des produits éligibles aux labels les aux labels les plus exigeants. Ces objectifs, certes ambitieux, se heurtent à une double réalité : à un manque de disponibilité de la matière première française pour répondre au choc de la demande-

à court terme. Pis, il risque de se traduire par une augmentation du nombre de produits importés. La seconde posture est celle qu'a choisie la commission des affaires économiques, qui considère que la priorité absolue est de s'attaquer à très court terme à la part des produits importés dans notre restauration collective, pour atteindre à la fois les objectifs de la loi Climat et ceux de la loi Égalim pour une alimentation saine et durable. Une telle option implique d'élargir la liste des produits français à privilégier dans les cantines à d'autres produits de nos régions respectueux de l'environnement et d'un cahier des charges. C'est ainsi que la commission a inséré dans la liste des produits à privilégier par les gestionnaires les produits locaux et les produits sous certification de conformité, dans la mesure où ils répondent à un cahier des charges exigeant. Les deux options, vous l'avez compris, ne sont pas compatibles à court terme. Rehausser les objectifs ou restreindre la liste, comme les auteurs de certains amendements le proposent, impliquera une équation impossible à résoudre à résoudre pour nos gestionnaires, qui recourront alors à des produits importés, disponibles, éligibles et moins chers. C'est pourquoi je vous proposerai une solution visant à faire de la lutte contre les produits importés la priorité pour favoriser les produits français, y compris, bien sûr, les produits sous SIQO, qui bénéficieront bien évidemment d'une explosion du marché avec le déploiement du dispositif à la restauration collective privée et aux services de l'État. La parole

Malheureusement, l'examen en commission des affaires économiques du Sénat a conduit à amoindrir les objectifs d'un article déjà peu ambitieux. Pourtant, il est aujourd'hui indispensable, pour des raisons environnementales, mais aussi pour la qualité des repas, que ce soit sur le plan nutritif et pour la santé de nos concitoyens, d'améliorer significativement l'encadrement des produits servis dans la restauration collective. Ainsi, il n'est plus acceptable de retrouver dans la liste des produits de qualité autorisés des produits dits HVE 2, qui ne correspondent plus aux critères définis, aux côtés de produits ayant une certification de niveau 3, qui répondent bien plus nettement aux objectifs environnementaux et sanitaires.

n'oublions pas que les agriculteurs ont fait des efforts pour atteindre les premiers niveaux de certification. Toutefois, la responsabilité du législateur est de toujours s'orienter vers la meilleure perspective pour l'intérêt général. Mes chers collègues, dans le cadre de l'examen de cet article 60, soyons ambitieux, en ne prenant en compte que le niveau 3 de la certification haute valeur environnementale pour les 50 % de produits

Nous en arrivons au sujet de la qualité de l'alimentation dans la restauration collective. Les amendements tendant à définir la qualité sont intéressants, car ils dessinent en creux le modèle agricole que nous souhaitons développer. En effet, cet article, comme d'autres dans le projet de loi, fait craindre des reculs en matière de développement de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est reconnue comme un modèle performant sur les plans tant économique

et diversifiée. Pourtant, si nous retraçons l'histoire de ces dernières années- fin du financement national de l'aide au maintien ; mise en place d'un crédit d'impôt pour la HVE

Aujourd'hui, le cahier des charges de la HVE n'est pas suffisant, comme le montre une note de l'OFB, que vous n'avez toujours pas rendue publique, nous vous avons saisi par un courrier il y a peu de temps de cette demande. Pour remédier à ce très mauvais signal, nous proposons donc plusieurs amendements visant à renforcer la part du bio dans la définition de la qualité et à limiter celle de la HVE, afin de faire preuve de cohérence et de permettre une réelle transition alimentaire. Les agriculteurs biologiques ont besoin d'être soutenus ; ils ont aussi besoin d'être rassurés. Monsieur le ministre, je tiens à vous dire que les propos que vous avez

tant qu'une réforme du cahier des charges de la HVE n'aura pas abouti. En effet, cette certification repose sur un cahier des charges incohérent, notamment pour les systèmes d'élevage, qui ne garantit pas aujourd'hui la qualité des produits, comme l'ont démontré un récent rapport de l'Iddri rapport de l'Iddri et une note de l'Office français de la biodiversité, dont nous attendons toujours la publication. Si un label environnemental intermédiaire entre le bio et l'agriculture conventionnelle pouvait présenter un intérêt, et si la HVE était ce label, il faudrait pour autant que le cahier des charges soit cohérent. L'idée n'est pas ici de dire que seuls les produits bio présentent un intérêt. D'autres dispositifs permettent d'avancer, notamment notamment les systèmes herbagers, le porc sur paille, le travail sur les rotations et sur les haies et les surfaces d'intérêt écologique. Mais, aujourd'hui, la HVE n'apporte pas de garanties. Une réforme de la certification est nécessaire avant que d'en faire un outil efficace de politique publique. Elle est d'ailleurs en cours et devrait aboutir en janvier 2023, d'après les échos que j'ai entendus, pour modifier en profondeur le cahier des charges. M. le ministre pourra peut-être nous apporter des précisions à ce sujet. Aussi, il est proposé, par cet amendement, de supprimer la possibilité pour les produits issus du plus haut niveau de la certification HVE d'entrer dans les 50 % de qualité en restauration collective jusqu'à la date de 2023, le temps de prévoir une évolution cohérente du cahier des charges de la HVE. Il est en effet incohérent d'orienter les soutiens publics vers la HVE tant que sa performance environnementale n'est pas démontrée et alors qu'une réforme majeure de son cahier des charges est en cours. Cette catégorie est en effet actuellement utilisée pour détourner la notion de qualité alimentaire des produits de la restauration collective. À titre d'exemple, la charte EVA, qui certifie aujourd'hui la quasi-totalité de la volaille standard française, vient d'obtenir la certification environnementale de niveau 2. Ainsi, ces produits, qui correspondent à un modèle d'élevage intensif, peuvent intégrer les 50 % de produits durables

dans le cadre des dispositions de la loi Égalim. Nous sommes très attachés à la préservation et à la défense des produits sous signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine. Ces SIQO répondent à de hauts niveaux de qualité alimentaire et sont identifiés et appréciés par les consommateurs. Or la rédaction actuelle du code rural, même en prenant en compte les modifications opérées par le présent projet de loi, met en place une concurrence déloyale pour ces produits au profit d'autres produits ne présentant pas nécessairement les mêmes gages de qualité. Afin d'accorder aux produits sous SIQO la place qui devrait être la leur, sans remettre en cause les objectifs de montée en gamme déjà inscrits dans la loi, cet amendement vise à porter de 50 % à 60 la part des produits de qualité servis dans les restaurants collectifs d'ici à 2022, de prévoir que 20 % devront être sous SIQO et de maintenir l'objectif de 20 % des produits issus de l'agriculture biologique. Je précise que nous considérons la

présenter l'amendement n° 316 rectifié. L'une des conclusions des États généraux de l'alimentation menés en 2018 était de permettre l'accès à tous, notamment dans le cadre de la restauration collective publique, à une alimentation de qualité, saine, durable et d'origine locale, en particulier à des produits locaux ou sous signes officiels de qualité. Tel qu'il est rédigé, cet article permet à une grande partie de la production standard française d'entrer dans cet objectif, à la place des produits locaux sous signes officiels de qualité. C'est une bonne chose pour favoriser la production française, mais cela aura clairement un impact négatif pour les produits sous signes officiels d'identification de la qualité et de l'origine dans la restauration collective, car ils sont de fait plus chers que la production standard.

de produit représente tous les volumes de volailles achetés par le secteur de la restauration collective, puisqu'il est moins cher que les volailles fermières label rouge, IGP ou bio. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Un référentiel belge concernant des légumes a également été reconnu en certification environnementale de niveau 2.

à rehausser les seuils à atteindre. Je le rappelle, la priorité à court terme est bien de lutter contre les produits importés, et non de durcir les seuils à atteindre pour une liste de produits trop restrictive, évinçant au final bon nombre de produits français. Il est important de ne pas envoyer de signaux contradictoires aux gestionnaires et de maintenir les objectifs déjà ambitieux que nous avons fixés il y a seulement deux ans. On estime que les objectifs à atteindre- 50 % et 20 % -sont aujourd'hui à 15 % et 7 7 %. Nous en sommes à rehausser les objectifs, alors que nous n'arrivons même pas à atteindre les cibles fixées depuis deux ans ! Proposons donc plutôt des solutions opérationnelles aux gestionnaires en élargissant la liste et en arrêtant de modifier sans cesse les objectifs fixés par le législateur à chaque loi. Les amendements n 1208 rectifié, 1905 et 1628 changent les règles du jeu une fois encore, alors même que les gestionnaires viennent seulement de se structurer. L'avis est donc défavorable. Les amendements n 316 rectifié bis et 1146 sont au final contradictoires et difficilement lisibles quelle est la différence entre un objectif de 50 % de produits Égalim, à savoir majoritairement des produits bio et SIQO, et le taux préférentiel proposé de 30 % pour des SIQO qui, eux-mêmes, intègrent des bio ? Franchement, cela devient un vrai casse-tête pour les gestionnaires ! Je voudrais vraiment appeler l'attention de mes collègues sur le fait que ces amendements sont très restrictifs : leur adoption conduirait, au final, à évincer nos productions françaises, au bénéfice de produits importés moins chers

il faut arrêter de dire que c'est l'État qui fait de la surtransposition. Ce n'est pas vrai ! Peut-être qu'il en fait ici ou là, mais de nombreuses surtranspositions sont votées dans les hémicycles

dont 50 % de bio. Nous sommes presque en 2022, date fixée pour l'atteinte des objectifs d'intégration de bio et de qualité dans la restauration collective Il faut non pas en rester là- nous n'avons d'ailleurs pas encore atteint ces objectifs -, mais s'inscrire dans une démarche d'amélioration constante, en phase avec les attentes sociétales sur la qualité et la relocalisation de l'alimentation, ainsi qu'avec la protection de l'environnement et l'amélioration de la rémunération des agriculteurs. Les objectifs de montée en gamme sur les signes de qualité, travaillés lors des États généraux de l'alimentation, doivent être accompagnés par un développement de l'offre, notamment la restauration collective.

parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier. La pêche est un sujet de tension écologique extrêmement important pour nos environnements marins. Il est urgent de faire évoluer notre consommation de produits de la mer vers des pratiques plus durables. Une action forte sur la consommation de produits de la mer dans la restauration collective est susceptible d'engendrer une réduction significative de notre impact marin. Cependant, l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est très peu contraignant en termes de consommation de produits de la mer. Nous devons noter que rien n'impose que des produits de la mer soient inclus dans les 50 % de produits spécifiés. Nous observons d'ailleurs que, parmi tous les produits servis dans ces établissements, les produits de la mer sont les bons perdants en termes de labellisation durable, ce qui confirme l'intérêt de renforcer la contrainte prévue dans l'article en question.

je ne crois pas que prévoir une sous-catégorie soit une bonne solution : cela risque, une fois encore, de virer au casse-tête pour nos gestionnaires. J'ajoute que l'écolabel l'écolabel visé ne concerne qu'une poignée de produits et qu'il n'inclut pas les produits de la pêche label rouge. En pratique, il sera impossible d'atteindre le taux visé. En outre, l'amendement est quasi satisfait, puisque l'article prévoit, un peu plus loin, qu'il est obligatoire pour la restauration collective que les viandes et les poissons, avec les critères déjà prévus par la loi, représentent 60 % des taux d'approvisionnement globaux, y compris les SIQO.

Ces alinéas incluent, dans la liste des produits de qualité à proposer dans la restauration collective, les produits « dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement » des circuits courts et les produits locaux. Nous sommes très attachés, bien entendu, au développement des circuits courts et aux produits locaux- la multiplication de nos initiatives et amendements sur ce sujet le démontre -, mais nous estimons qu'il n'existe pas nécessairement de lien entre circuits courts et qualité de la production. Or l'utilisation de l'expression « fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement » pourrait laisser la place à une large interprétation qui ne correspondrait pas à l'esprit de la loi. Il ne faudrait pas envoyer un mauvais message à des filières qui répondent actuellement à des cahiers des charges très stricts pour bénéficier d'un signe de qualité reconnaissable et reconnu. C'est pourquoi, au vu du flou de la rédaction de l'alinéa 5, nous en proposons la suppression. Quel est l'avis de économiques ? Nous avons effectivement mis en place un dispositif qui permet aux produits locaux et aux circuits courts d'être pris en compte et privilégiés dans la restauration collective. C'est, je le pense, une oeuvre utile essentielle pour atteindre les objectifs d'Égalim et qui est attendue par nos gestionnaires et les usagers pour mieux localiser notre alimentation en utilisant le levier de la restauration collective et pour structurer- on sait combien c'est important -les filières locales. Une alimentation plus locale, c'est une alimentation qui répond à l'objectif de ce projet de loi, c'est-à-dire qui a une empreinte carbone réduite. J'ajoute que nous avons précisé, mon cher collègue, un critère de qualité et un critère environnemental, qui permettent à ces produits d'entrer pleinement dans les 50 % d'Égalim. L'avis est défavorable. Quel est l'avis

officiels de qualité et d'origine : leurs cahiers des charges encadrent précisément un certain nombre d'opérations concernant le produit pour que celui-ci bénéficie du logo label rouge ou IGP, jusqu'à la transformation et le conditionnement. Par exemple, la viande crue bénéficie du label rouge, mais pas les produits précuits et prétranchés, qui intéressent la restauration collective, car ces modes de présentation ne sont pas prévus dans les cahiers des charges. Aussi, pour

des marques Valeurs parc naturel régional et Esprit parc national répondent totalement aux objectifs de l'article 24 de la loi Égalim. Nous estimons anormal, tant pour les producteurs qui se sont inscrits dans les démarches de ces marques que pour les élus locaux qui font vivre les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux, que ces produits soient exclus des 50 % de produits obligatoires de la restauration collective d'ici à 2022.

Elles sont porteuses des valeurs de ces aires protégées que sont les parcs naturels régionaux et les parcs nationaux et distinguent des produits conciliant aspects écologiques, économiques et sociaux. Quel est l'avis de la commission

Si nous sommes très attachés au développement du niveau de certification 3, qui répond à de véritables critères de qualité, nous nourrissons des réserves sur les niveaux de certification environnementale inférieurs, non pas dans l'absolu, mais parce qu'ils s'inscrivent dans une trajectoire de progrès vers le niveau 3. C'est pourquoi, par cet amendement, nous proposons que seul le niveau 3 de la certification HVE puisse entrer dans les 50 % de produits de qualité en restauration collective. Bien évidemment, le niveau HVE 2 pourra toujours être servi dans la restauration collective, mais au titre des autres 50 % que nous pourrions qualifier de standards.

repli vise à rétablir les deux alinéas supprimés en commission concernant l'avancement du calendrier autorisant uniquement les produits HVE 3, tout en étant plus ambitieux que le texte issu de l'Assemblée nationale. Ainsi, nous proposons de fixer à 2025 la date à partir de laquelle seuls les produits certifiés HVE 3 seront comptabilisés dans la liste des 50 % de produits durables.

tenter de vous convaincre. Cet amendement vise à rétablir les deux alinéas supprimés en commission concernant l'avancement du calendrier autorisant uniquement les produits HVE 3, en retenant cette fois la rédaction de l'Assemblée nationale, à savoir 2027. La parole est à Mme Patricia Schillinger, L'article 60 étend à la restauration collective privée les dispositions de la loi Égalim prévoyant l'obligation de proposer une part de produits durables et de qualité à hauteur d'au moins 50 %, dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique. La commission a choisi de revenir sur une proposition de la rapporteure de l'Assemblée nationale, qui a souhaité anticiper la fin de la tolérance pour les produits sous certification environnementale de niveau 2. Notre amendement tend à accélérer la transition vers le niveau 3, qui vise la haute valeur environnementale, en modifiant la date butoir pour choisir le 31 décembre 2026. Nous pensons que l'échéance doit être compatible avec la réalité ; or de nombreuses exploitations sont entrées

Avec cet amendement, nous choisissons d'accompagner l'engagement des producteurs, déjà nombreux à s'être inscrits dans cette démarche de certification, et d'inciter à produire toujours mieux avec des produits de meilleure qualité.

La commission des affaires économiques du Sénat a fait le choix d'ajouter les produits bénéficiant d'une démarche de certification de conformité des produits (CCP) à la liste des produits compris dans les 50 % de produits durables et de qualité à intégrer en restauration collective. Pourtant, le certificat de conformité n'est pas une garantie suffisante de qualité. De ce fait, cette disposition n'est pas cohérente avec l'esprit initial de la mesure, à savoir favoriser la qualité alimentaire et environnementale en restauration collective.

Il est donc proposé de revenir sur cette disposition adoptée en commission et de supprimer une telle mention dans la liste des produits de qualité définie à l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime.

auront un cahier des charges qui devra être contrôlé et validé par l'État et qu'il devra comporter des mesures environnementales et de qualité suffisantes. Les paramètres de qualité

des exploitations, l'un des principaux indicateurs de la « durabilité » des systèmes d'élevage. Dans l'objectif de faciliter l'approvisionnement en viandes durables et de lutter contre les viandes d'importation en restauration collective- elles représentent 48 % des approvisionnements -, il semble pertinent d'intégrer ce critère à la liste fixée par la loi Égalim pour accéder à l'objectif de 50 % d'approvisionnement en produits durables.

n° 996 rectifié. En France, l'autonomie fourragère des exploitations d'élevage de ruminants fait partie des spécificités et des principaux atouts de notre modèle en moyenne, 60 % de l'alimentation fournie aux bovins est produite par l'éleveur sur son exploitation. Ce taux s'élève même à 80 % pour les cheptels allaitants. C'est pour valoriser cet atout du modèle d'élevage français et engager les éleveurs sur la voie d'une amélioration de leurs pratiques sur ce plan que le présent amendement vise à intégrer ce critère d'autonomie des exploitations dans la liste des critères d'éligibilité aux 50 %, fixés par la loi Égalim, d'approvisionnement en produits durables des restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge. La parole est à M.

Le présent projet de loi vise à rendre cohérente la définition de la qualité alimentaire telle qu'elle est prévue par la loi Égalim pour l'approvisionnement en produits durables et de qualité en restauration collective. collective. Aujourd'hui, l'objectif de cette disposition est détourné, et certaines productions d'élevage les plus intensives peuvent y être intégrées la certification environnementale de niveau 2, dont le cahier des charges est inopérant concernant l'élevage. À titre d'exemple, la charte EVA, qui certifie aujourd'hui la quasi-totalité des volailles standards françaises, vient d'obtenir la certification environnementale de niveau 2 par un arrêté du 25 janvier 2021. Ainsi, ces produits peuvent désormais intégrer les 50 % de produits durables en restauration collective. L'amendement vise à éviter ces dérives et à exclure les et à exclure les productions d'élevage qui ne bénéficient pas d'une mention valorisante de qualité reconnue au niveau européen par le règlement de commercialisation des volailles, ainsi que les productions issues de poules pondeuses en cage et d'élevage soumis à autorisation environnementale. Il apparaît essentiel, au-delà de l'extension de l'article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime à la restauration collective privée, de favoriser les élevages français répondant à des normes élevées de qualité, de bien-être animal et de respect de l'environnement.

l'ensemble des produits est comptabilisé, et il est fort probable que certaines filières, à commencer par celle des fruits et légumes, seront davantage mobilisées pour atteindre cet objectif. Le présent amendement vise donc à s'assurer de la diversification des produits permettant d'atteindre le 20 % en bio, en précisant que, pour les produits carnés et de la mer, 20 % en valeur devront être issus de l'agriculture biologique.

celle évoquée à l'Assemblée nationale pour prévoir une nouvelle obligation de proposer un menu végétarien quotidien alternatif dans les restaurants collectifs gérés par l'État, entreprises publiques nationales, il est ici proposé en contrepartie de concrétiser cette exemplarité par un objectif d'approvisionnement à 100

Cet amendement vise à faire de l'État, de ses établissements et des entreprises publiques nationales des exemples dans ce domaine, en leur demandant d'atteindre des objectifs plus ambitieux. Cette logique d'exemplarité se concrétisera par un objectif de 80 % dès 2024, contre 60 % pour les autres gestionnaires, et 100 % en 2027.

L'exemplarité des pouvoirs publics dans ce domaine est une nécessité. Tel est l'objet du présent amendement. Toutefois, le taux de 100 % que nous venons de défendre pourrait être dissuasif et générer des inquiétudes dans sa mise en oeuvre. C'est pourquoi cet amendement vise à proposer un taux de 80 %, plus ambitieux que celui de 60 % qui sera appliqué à l'ensemble de la restauration collective, publique et privée, en 2024.

Jacquin. Cet amendement vise à privilégier un approvisionnement local dans la part de produits durables et de qualité servis en restauration collective.

de rendre un rapport sur la mise en oeuvre des objectifs d'approvisionnement en produits durables et de qualité dès le 1 janvier 2022, date même de l'entrée même de l'entrée en vigueur de ces objectifs. Les opérateurs ont engagé des démarches pour permettre le suivi précis de l'ensemble des produits entrant dans ces objectifs, mais ce suivi demande du temps avant d'être opérationnel. Il est aussi proposé de remettre chaque année

Cet amendement vise à préciser que ce bilan statistique annuel évalue aussi la part des produits de qualité issus des circuits courts et de ceux d'origine française. Comme vous avez pu le constater, nous sommes favorables au maintien d'un niveau de qualité important pour les produits servis en restauration collective. Nous espérons que cet objectif permettra de structurer une offre locale ou nationale. C'est pourquoi nous pensons important que le bilan annuel se penche également sur ces deux dimensions afin d'évaluer l'évolution de l'origine de l'approvisionnement par les gestionnaires de restaurants collectifs. Si la réalisation des objectifs de la loi Égalim revenait à importer davantage de produits étrangers, nous serions ainsi mieux à même de tirer la sonnette d'alarme et de tenter de rectifier le tir pour que la loi bénéficie avant tout à nos producteurs.

La question de la qualité de notre alimentation et des repas servis dans la restauration collective est liée à celle de la relocalisation des productions agricoles. Pour nous, il s'agit de deux volets qui doivent être traités de façon conjointe. de façon conjointe. Afin de répondre aux enjeux climatiques liés à l'élevage, de faire évoluer qualitativement la consommation de viande servie dans la restauration collective publique et d'assurer à nos éleveurs des débouchés pour leurs productions de qualité, nous souhaitons renforcer, d'ici au 1 janvier 2023, les obligations attachées aux viandes de boeuf, de veau, d'agneau ou de volaille servies dans les restaurants collectifs dont les personnes publiques ont la charge. Nous proposons ainsi de fixer un objectif spécifique d'approvisionnement en viande locale et durable, sur le modèle de l'objectif multi-produits fixé par la loi Égalim. Quel

J'ajoute qu'à l'article 60 une rédaction alternative, mais quasiment identique, a prévu un objectif de viandes répondant à ces critères dans la restauration collective, comme dans la restauration privée, à hauteur de 60 %, en prévoyant des démarches certifiées

L'article 6 de l'ordonnance n° 2019-1110 du 30 octobre 2019 a, quant à lui, rendu possible cette adaptation au plus tard le 14 avril 2020. Or aucun décret n'a été publié. Au 1 janvier 2022, ce sont donc les obligations actuellement définies dans la loi qui s'appliqueront partout. Du fait de la faible offre locale de produits issus de l'agriculture biologique dans ces territoires, l'obligation de 20 % de produits biologiques se traduira mécaniquement par des importations de ces produits,

Compte tenu de la situation particulière des agricultures ultramarines, la loi Égalim avait effectivement prévu qu'un décret puisse adapter les seuils de produits à privilégier dans la liste, afin d'éviter des importations trop importantes.

en proposant que la convention passée entre le directeur de l'établissement scolaire, collège ou lycée, et le président du conseil départemental ou du conseil régional comprenne un volet relatif à la restauration scolaire.

À l'heure actuelle, les départements ou les régions souhaitant prendre des initiatives en matière de restauration scolaire se trouvent en effet démunis, faute d'un réel pouvoir sur ces gestionnaires. Alors que le projet de loi dit 3DS permettra d'aborder ce renforcement du pouvoir d'instruction des présidents de conseil départemental ou de conseil régional sur les gestionnaires des collèges et lycées,

Dans un rapport d'évaluation de 2019, le CGAAER estime que la mise en oeuvre de la loi Égalim dans la restauration collective induit un surcoût compris entre 0,10 euro et 0,42 euro. Si ce rapport précise, toutefois, que ce surcoût pourrait être compensé par la lutte contre le gaspillage alimentaire, une meilleure organisation de la programmation de l'approvisionnement ou un grammage mieux adapté aux besoins,

de remettre, dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport au Parlement sur l'opportunité de mettre en place un fonds d'aide à la transition alimentaire de la restauration collective publique.

à préciser que les chèques alimentaires doivent non seulement concerner la qualité nutritionnelle des produits, mais aussi garantir la durabilité des conditions de production des produits vers lesquels ils sont fléchés. La proposition de la Convention citoyenne pour le climat était de de produits durables : « Mettre en place des chèques alimentaires pour les plus démunis, à utiliser dans les AMAP ou pour des produits bio. » En qualifiant le chèque alimentaire seulement de nutritionnel, sans référence à la durabilité et à la qualité de l'alimentation,

On donne aussi potentiellement une image stigmatisante des bénéficiaires de l'aide alimentaire, en estimant que le chèque doit leur apprendre à manger sainement, c'est-à-dire uniquement des produits avec une qualité nutritionnelle. Cela ne nous paraît pas pas souhaitable. Sans préjuger de manière trop catégorique le dispositif, qui, on l'a compris, est encore en cours d'élaboration, il semble essentiel d'apporter des garanties sur la qualité environnementale de l'alimentation proposée dans le cadre du chèque alimentaire.

Olivier Jacquin. Nous proposons de compléter le rapport gouvernemental prévu dans cet article par l'examen d'une piste supplémentaire pour répondre à l'urgence de la précarité alimentaire et au défi de la démocratisation de l'accès à une alimentation durable. L'idée est celle d'un « chèque déjeuner pour tous tous », sur le même principe que le titre-restaurant, cofinancé par l'entreprise, l'employeur bénéficiant d'une réduction de charges sociales. L'idée est aussi d'étendre ce dispositif à tous les Français pour ne pas stigmatiser les plus précaires. Un mécanisme général de grands principes

faciale, la durée et le financement de ce dispositif. Le chèque alimentaire a pour objectif de permettre le développement de la consommation de produits agricoles et agroalimentaires de qualité par l'ensemble de ses bénéficiaires. Il s'agit non seulement de réduire les inégalités alimentaires et nutritionnelles, mais aussi d'accompagner la structuration de filières agricoles. Dès lors, il ne nous semble pas opportun de restreindre son bénéfice aux seuls produits frais, les produits transformés pouvant également convenir. C'est la raison pour laquelle nous proposons la suppression de cette mention au titre des objectifs visés par ce rapport.

En favorisant l'accès à des produits sains et durables, les chèques alimentaires peuvent réduire le cumul des inégalités sociales et de santé. En cette période de crise sanitaire, ils représentent également un soutien nécessaire pour les personnes qui vivent dans la précarité. Cet amendement vise à compléter le rapport proposé pour s'assurer que ces chèques alimentaires répondent aux besoins des usagers, tout en constituant un levier de développement d'une production agricole locale, écologique, de qualité, et de construction d'une démocratie alimentaire. Pour cela, nous proposons que le rapport étudie la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation associant l'ensemble des acteurs, en particulier les usagers. usagers. Nous prévoyons également un travail sur les modalités de distribution des produits liés à ces chèques, en particulier dans les zones où les points de distribution sont absents ou insuffisants. effet, il est aussi essentiel d'assurer l'accessibilité physique à une offre alimentaire durable et de qualité, aujourd'hui peu présente dans les zones les plus défavorisées. Le rapport Le rapport pourrait ainsi étudier les mécanismes de soutien à l'agriculture urbaine, l'installation de marchés ou de magasins de producteurs, d'épiceries solidaires, de groupements d'achat, d'AMAP solidaires dans les quartiers défavorisés, par exemple grâce à un fonds dédié. Nous demandons par ailleurs que le rapport fournisse un travail sur l'offre alimentaire de qualité durable, afin d'assurer l'approvisionnement des denrées alimentaires choisies par les utilisateurs Ce dispositif doit en effet relier alimentation et agriculture, politique alimentaire et politique agricole. Enfin, nous souhaitons que le rapport étudie des mécanismes d'accompagnement et de pédagogie, de partage de savoirs et d'informations sur l'alimentation saine, locale et durable, ainsi que sur les systèmes agricoles, afin, notamment, de contribuer à relier citoyens et agriculteurs. Il est important de préciser le contenu de ce rapport sur lequel nous avons, pour l'instant, peu de garanties.

La crise sanitaire a entraîné un renforcement de la précarité économique et alimentaire. Dans un contexte d'urgence, les chèques alimentaires constituent une avancée notable, et nous serons très vigilants sur la mise en oeuvre du dispositif, pour l'instant encore peu concret. Il nous faut articuler dès aujourd'hui des réponses beaucoup plus structurelles pour assurer un vrai droit à l'alimentation. Le système actuel d'aide alimentaire présente en effet des lacunes. Il ne fait notamment pas le lien entre précarité alimentaire, santé publique, transition agroécologique et rémunération juste des producteurs. Or, aujourd'hui, l'accès financier aux produits de qualité et durables est difficile pour les plus précaires. Afin de rendre l'alimentation de qualité accessible à tous, tout en rémunérant les producteurs, il faut mener une réflexion sur ces enjeux interdépendants. L'évolution vers une sécurité sociale de l'alimentation durable, conçue comme une politique publique transversale, permettrait de répondre à ces enjeux économiques, sociaux et environnementaux en versant un montant fixe tous les mois à un public ciblé, voire progressivement élargi, la sécurité sociale. Ce montant serait à dépenser dans les établissements conventionnés et pour des produits conventionnés. Il s'agirait d'un mécanisme inclusif, qui permettrait d'accélérer la transition agroécologique, tout en travaillant sur une rémunération équitable des producteurs. Certes, le coût de cette mesure est élevé, mais il est à amortir sur le long terme grâce aux économies sur les

d'une utopie diront certains, mais une utopie nécessaire, comme l'était la sécurité sociale à l'origine. Un rapport parlementaire sur le sujet, prévoyant notamment les modalités d'une concertation sur cette idée, serait une première étape pour faire avancer cette question du droit à l'alimentation.

effectivement d'accompagner les personnes de manière régulière, sans mettre en action une cohorte d'acteurs sociaux, serait peut-être beaucoup plus équilibré que les systèmes actuels. C'est une orientation politique particulièrement intéressante à travailler.

Pour sa part, la commission des affaires économiques considère que le problème de la précarité alimentaire nécessite d'abord des solutions concrètes, comme celles que nous venons d'évoquer : un chèque alimentaire bien ciblé ; une aide alimentaire prenant mieux en compte les impératifs de qualité, tout en maintenant un volume suffisant. L'avis est donc plutôt défavorable.

Dans le cadre de la lutte contre la précarité alimentaire et de l'aide aux plus démunis, l'urgence à nourrir prime. Cependant, la qualité ne peut pas pour autant être négligée. l'on rogne sur la qualité au profit des prix les plus bas, sans contrôle suffisant, le risque demeure de voir ressurgir une situation similaire à celle de 2019, lorsqu'a éclaté le scandale des steaks hachés frauduleux distribués aux associations d'aide alimentaire dans le cadre du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD). L'excellent rapport sénatorial qui avait été réalisé sur cet épisode avait d'ailleurs conclu à la nécessité d'imposer, dans les appels d'offres, des critères de qualité sur les produits, des critères à concilier, bien évidemment, avec les quantités nécessaires dans le cadre de l'enveloppe allouée. Nous y proposions également des pistes de mise en oeuvre, avec, notamment, de meilleures méthodes d'allotissement, un rythme pluriannuel et l'expérimentation d'une séparation des appels d'offres pour la production de denrées et pour la logistique. Cet amendement vise à préciser la prise en compte de critères de qualité des denrées dans la mesure du possible, au vu des quantités nécessaires, dans les objectifs de la politique d'aide alimentaire.

Cet amendement a pour objet de renforcer l'inscription dans la loi de l'objectif de la stratégie nationale pour le développement des protéines végétales, qui concerne les légumineuses, à savoir 8 % de la SAU en 2030, adopté par la commission des affaires économiques, en lui ajoutant un objectif complémentaire, à l'horizon de 2050, de 15 % de la SAU. Les filières sont aujourd'hui mobilisées pour développer les légumineuses, à la fois pour l'alimentation humaine Pour accélérer ce mouvement, il est important pour les auteurs du présent amendement de fixer des objectifs clairs dans la loi, y compris à l'horizon de 2050. Alors que le présent projet de loi prévoit, à l'article 62, une réduction des engrais azotés, et que l'article 59 que nous venons de voter vise à introduire des protéines végétales en restauration collective, acter un signal fort sur les légumineuses semble essentiel. Cet amendement vise également à préciser que les cultures de légumineuses doivent être diversifiées, afin de garantir l'efficacité de ces cultures pour la réduction des intrants et la transition écologique de l'agriculture et de l'alimentation.

Cet amendement vise à inscrire dans la loi les objectifs du en termes de développement de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, on l'a dit, est un levier essentiel pour la transition agricole. Les objectifs fixés dans la loi sur l'agriculture, à savoir 15 % des surfaces en bio en 2022, vont bientôt arriver à échéance, et on est loin du compte. Plutôt que d'en rester à ces objectifs, il convient de s'inscrire dans une progression continue du développement de l'agriculture biologique en actant les objectifs du, à savoir utile) en bio en 2030, afin d'envoyer un signal fort à l'ensemble des acteurs sur cette orientation. Des manifestations d'agriculteurs bio ont eu lieu un peu partout sur le territoire, car ils ressentent un véritable manque de soutien après la fin du financement national de l'aide au maintien et la baisse du financement de la PAC, et ce alors qu'ils rendent des services à la collectivité pour la qualité de l'air et contribuent à toutes les externalités positives. Le présent amendement vise à réaffirmer que ce modèle est un outil essentiel de la transition agroécologique, de l'atteinte des objectifs climatiques et de la réduction des pollutions atmosphériques, et à aligner ainsi la France sur les objectifs européens en la matière. Quel est l'avis de la commission

tenable, et qui mobilise toutes les forces en présence. Il devra notamment s'appuyer sur une étude d'impact pour mesurer les effets de telle ou telle décision. Au niveau européen, cet objectif fait aussi l'objet de débats. Il nous semble donc trop tôt pour l'inscrire en dur dans la loi.

On peut dire que ce n'est pas assez ; moi-même, je pense qu'il faut aller encore plus loin. Mais voilà tout de même ce que nous sommes en train de réaliser

amendement vise à introduire dans les objectifs-cadres de notre politique en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, définie à l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, le fait de reconnaître et de mieux valoriser les externalités positives de l'agriculture, notamment en matière de services environnementaux et d'aménagement du territoire. Les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain sont très attachés à la reconnaissance des externalités positives de l'agriculture, notamment à la valorisation des paiements pour services environnementaux en agriculture, dont l'intérêt est aujourd'hui reconnu par tous. Les PSE sont en effet un outil pouvant allier une nécessité économique à une attente sociétale en valorisant les externalités positives de l'agriculture, c'est-à-dire les effets positifs de l'agriculture sur les écosystèmes qui peuvent être engendrés par des modes de production ou des pratiques adaptés. Nous estimons que les PSE permettent de sortir de la seule logique, au demeurant toujours nécessaire, de compensation des surcoûts ou des manques à gagner, qui domine actuellement dans les politiques agricoles, et d'encourager, en les rémunérant dans la durée et si possible hors du cadre de la PAC, les éléments de préservation et de valorisation de la biodiversité, ainsi que les pratiques qui permettent d'améliorer la santé et l'efficacité agronomique, climatique et environnementale des écosystèmes. Dès 2018, je le rappelle, nous avions porté en séance publique une proposition de résolution en faveur de leur généralisation. Au vu de l'intérêt stratégique, environnemental, économique, et parfois culturel, de la valorisation des externalités positives de notre agriculture, notamment des PSE, nous estimons qu'il est désormais temps de les reconnaître à l'article L. 1 du code rural pour consacrer dans la loi leur existence et y inscrire la nécessité de les développer. ? L'oubliée de ce projet de loi est effectivement la valorisation des externalités positives de l'agriculture, comme celle de la forêt d'ailleurs. Tout se passe comme si nos agriculteurs étaient un fardeau environnemental. On oublie trop souvent l'ensemble des services sociaux et environnementaux qu'ils rendent à nos concitoyens en matière de stockage de carbone, de préservation de la biodiversité, d'aménagement du territoire et d'animation de la vie rurale. Ces externalités positives doivent être mieux valorisées. Nous partageons cet objectif. La commission

et de notre société en général. Dès 2018, nous défendions une proposition de résolution en ce sens. Quelques mois plus tard, dans le cadre du plan Biodiversité, 150 millions d'euros étaient mobilisés sur les programmes d'intervention des agences de l'eau pour valoriser ces pratiques. Si nous saluons cette avancée, nous estimons néanmoins qu'une massification des efforts est plus que jamais nécessaire au vu des défis environnementaux, climatiques et économiques auxquels nous devons faire face. Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement la remise d'un rapport dressant un état des lieux de la mise en oeuvre des PSE en France, de l'identification des freins ou leviers dans ce domaine et de la mise en place d'une trajectoire de développement. Il s'agit d'avoir un point d'étape fiable de la situation actuelle pour savoir d'où nous partons, de nous fixer des objectifs que je souhaite ambitieux et de déterminer en conséquence les trajectoires à adopter et les outils à mettre en place pour les atteindre. Je sais que le Sénat n'aime pas trop les rapports, mais celui-ci présenterait un réel intérêt. Monsieur le ministre, je souhaite que le Gouvernement nous suive, dans le droit fil du vote de l'amendement précédent reconnaissant les externalités positives et les services environnementaux de l'agriculture.

amendement s'inscrit dans la continuité des précédents en faveur des PSE. Il vise à créer un nouvel article dans le Livre Préliminaire du code rural et de la pêche maritime, afin de préciser que les politiques en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt,

les auteurs de cet amendement proposent une définition du concept d'aménité rurale et les modalités générales pour les encourager l'État et les collectivités territoriales. Le projet de loi Climat met en avant le terme de résilience, mais ne le définit pas. Cet amendement vise à répondre à la nécessité d'identifier les aménités rurales comme un moyen, juridiquement fondé, de contribuer à la résilience de notre société, grâce à la ruralité.

que du maintien des prairies permanentes. Pour atteindre les objectifs de réduction d'émissions de CO2 dans le secteur agricole, la haie est un outil indispensable. Les haies permettent, à la fois, d'atteindre des objectifs climatiques le stockage de carbone, en plus de préserver les fonctionnalités du sol et les continuités écologiques, et de jouer localement un rôle paysager. Elles ont aussi un intérêt agronomique en abritant des auxiliaires de culture et en limitant la diffusion des pathogènes. Quand elles sont bien gérées, elles permettent le développement d'une ressource locale et durable de bois énergie, ce qui constitue une ressource supplémentaire pour les agriculteurs. Aujourd'hui encore, nous perdons chaque année

De même, les prairies permanentes constituent un puits de carbone naturel, en plus d'être un milieu essentiel pour la biodiversité. De nombreuses études et des outils diagnostics montrent que ces prairies sont un outil essentiel pour diminuer le bilan carbone et azoté des exploitations d'élevage de ruminants. Ainsi, cet amendement tend à fixer, parmi les objectifs de la politique en faveur de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche maritime, auxquels l'État se doit de veiller, un objectif de maintien des prairies permanentes, ainsi qu'un autre de préservation et de développement des haies

présenter l'amendement n° 33 rectifié. Cet amendement vise à ajouter deux impératifs pour parvenir à la souveraineté alimentaire de la France : garantir aux agriculteurs des prix rémunérateurs et les protéger de la concurrence déloyale de produits importés issus de systèmes ne respectant pas les normes de production imposées par la réglementation européenne. La parole est à Mme Dominique

Merci